en séance plénière, afin d'améliorer, pour les personnes handicapées, l'accessibilité au Palais du Luxembourg, à notre hémicycle et à ses tribunes. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'une campagne importante d'amélioration de l'accessibilité de nos locaux entamée depuis plusieurs années sur l'initiative des conseils de questure successifs. Je remercie tout particulièrement les questeurs de la réalisation effective de ce chantier.

communication du décret de M. le Président de la République en date du 28 juin 2017 portant convocation du Parlement en session extraordinaire.

Je souhaite la bienvenue à M. Michel Pélieu, qui a remplacé François Fortassin à compter du 16 mai 2017, et à M. Alain Poyart, qui a remplacé Patrick Masclet à compter du jeudi 15 juin 2017. Je salue le retour de nos quatre anciens collègues M. Jean-Vincent Placé, Mme Laurence Rossignol,

M. Gilbert-Luc Devinaz, qui a remplacé, en qualité de sénateur du Rhône, M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'intérieur, et à Mme Josiane Costes, qui a remplacé, en qualité de sénatrice du Cantal,

en application de l'article 5, alinéa 2, du règlement, la liste des sénateurs déclarant adhérer au groupe La République en marche, ainsi que la déclaration politique de ce nouveau groupe, qui compte vingt-huit membres. M. François Patriat, président de ce groupe, a également fait connaître que, en application de l'article 5 du règlement, le groupe La République en marche se déclare comme groupe minoritaire.

a en outre confirmé que son groupe se déclarait comme groupe minoritaire au sens de l'article 51-1 de la Constitution.

L'ordre du jour appelle la lecture de la déclaration de politique générale du Gouvernement. Au nom du Sénat,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est pour moi un plaisir et un honneur de lire aujourd'hui au Sénat la déclaration de politique générale que M. le Premier ministre,

je reste toujours optimiste. La vie m'a appris que, avec le temps, le progrès l'emportait toujours.

Ils ont été prononcés en 1995, mais ils sont éternels et ils sont ceux de la France. Ils disent ce qu'il faut d'effort et de courage pour que le progrès advienne. Ils disent aussi combien confiance et progrès ont partie liée. « Je veux, alors que je m'exprime depuis cette tribune devant la représentation nationale, après avoir cité Simone Veil, vous parler d'une autre femme, d'une femme qui, à la fin de l'été 2003, poussait les lourdes portes d'une grande école parisienne. Une jeune femme que rien ne prédestinait à entrer dans ce lieu. Une jeune femme qui a grandi en Seine-Saint-Denis, suivi une scolarité dans des établissements situés en quartiers d'éducation prioritaire, à Villetaneuse et à Saint-Ouen. Une jeune femme dont les parents, chauffeur-bagagiste et aide-soignante, ne s'attendaient pas à ce qu'elle accède à cette grande école parisienne, puis devienne avocate, puis travaille dans les cabinets les plus prestigieux, puis fonde son propre cabinet. Cette jeune femme siège aujourd'hui sur vos bancs. Sa réussite est le produit de son travail, de son engagement, de sa ténacité. Elle la doit aussi à la décision d'un responsable public, en l'occurrence le directeur de Sciences Po, qui avait, quelques années auparavant, bousculé son institution pour l'ouvrir à des formes d'excellence un peu moins classiques. Une politique publique, critiquée lorsqu'elle a été adoptée, copiée depuis et qui apparaît, quelques années après, grâce au travail et à l'effort de ceux qui en bénéficient, comme un modèle. Comme un progrès. « C'est long. C'est difficile. Mais ça a marché. Et pas seulement pour cette jeune fille : au moins deux d'entre vous ont bénéficié de cette politique publique audacieuse, dont un jeune homme de Saint-Laurent-du-Maroni, un des benjamins de cette assemblée, qui sera peut-être une de ces grandes figures que la Guyane offre parfois à notre pays. Des parcours individuels, certes, mais rendus possibles par une politique publique. « Ainsi va la République. Ou plutôt ainsi devrait-elle aller. Je regarde cette assemblée, je regarde ces bancs où je siégeais il y a quelques semaines encore. » N'importe quoi ! « Je vois un éleveur de la Creuse, agriculteur comme l'étaient son père, son grand-père et tellement d'autres avant lui, enraciné dans sa terre au point que le lieu-dit où il vit porte le nom de sa famille.

et a commandé une des compagnies de la Brigade franco-allemande. « Je vois un autre de vos benjamins, né au Rwanda quatre ans avant le génocide et recueilli par la République, qui lui a offert son meilleur visage et qui peut être fière de le voir aujourd'hui représenter la Nation. Je vois des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs, des scientifiques, des militants du monde associatif. Je vois même des matheux ! Des matheux qui, par leur talent et leur travail, constituent à la fois une fierté pour votre assemblée et une fierté pour la France. Je vois une assemblée rajeunie, féminisée, et largement renouvelée, puisque 430 d'entre vous font leurs premiers pas dans cette enceinte.

que se présente un gouvernement paritaire, lui aussi profondément renouvelé par la diversité de ses origines, professionnelles et politiques, et que le Président de la République m'a demandé de diriger. Je mesure cet honneur. « Je mesure la responsabilité, aussi, de la tâche qui est la mienne, et je l'aborde avec beaucoup d'humilité, avec une humilité d'autant plus grande que, pour préparer cette déclaration de politique générale, j'ai relu toutes celles de mes prédécesseurs. » Quelle depuis celle de Michel Debré, le 15 janvier 1959, jusqu'à celle de Bernard Cazeneuve, le 14 décembre dernier. Tous ces discours étaient inspirés par les convictions les plus sincères, par un patriotisme digne d'éloges et par le sens de l'État le plus élevé. Il faut avoir le courage de le dire, même si c'est à contre-courant des idées reçues : la France n'a jamais manqué de responsables politiques compétents et souvent d'une exceptionnelle qualité. Je sais d'ailleurs ce que je dois à l'un d'entre eux, Alain Juppé, et je voudrais ici lui rendre hommage. De tous ces discours, deux m'ont particulièrement marqué. « Je cite un extrait du premier ″De cette société bloquée, je retiens trois éléments essentiels : la fragilité de notre économie, le fonctionnement souvent défectueux de l'État, enfin, l'archaïsme et le conservatisme de nos structures sociales.″ « Ces mots sont d'une actualité criante ils ont été prononcés le 16 septembre 1969 par Jacques Chaban-Delmas, il y a

″Nos priorités ne sont pas celles d'une moitié de la France contre l'autre moitié, mais celles de tous les Français. Défaire ce que les autres ont fait, faire ce que d'autres déferont, voilà bien le type de politique dont les électeurs ne veulent plus. Nous ne demanderons à personne de nous rejoindre par intérêt ni de trahir ses convictions.″ Il s'agit des mots de Michel Rocard, le 29 juin 1988, il y a quand même presque trente Rocard, Chaban : deux personnalités éminentes, deux hommes d'État qui ont incarné deux courants essentiels de notre vie politique, le gaullisme et la social-démocratie deux hommes qui s'accordaient donc sur un constat et sur une méthode. « Et pourtant, le diagnostic posé il y a quarante-huit ans reste hélas valable la méthode proposée il y a trente ans demeure toujours une exigence, mais trop rarement une réalité. Et la France, à la différence de beaucoup de nations du monde, ne résout pas ses problèmes. En découle un sentiment mortifère où se mêlent désarroi, découragement, désenchantement et colère. Nous connaissons ce sentiment. Nous connaissons sa puissance. Nous le ressentons parfois nous-mêmes. Nos compatriotes l'ont exprimé, et fortement, lors de l'élection présidentielle, par un réflexe d'abstention ou un vote d'exaspération. Il faut comprendre ces angoisses, il faut entendre cette colère. « Mais nos compatriotes ont aussi exprimé un espoir formidable en portant Emmanuel Macron à la présidence de la République. Tandis que de grandes démocraties choisissaient le repli sur elles-mêmes, le dos tourné au monde, les Français, avec le Président de la République, ont préféré l'esprit d'ouverture et de conquête. « On leur proposait la nostalgie impuissante ; ils ont préféré le courage d'affronter l'avenir. Ils avaient à choisir entre la colère et la confiance ; ils ont exprimé leur colère, mais ils ont choisi l'optimisme et le rassemblement. Durant la campagne, depuis son élection et hier encore devant le Parlement réuni en Congrès, le Président de la République nous a montré le cap. J'en suis heureux : c'est bien souvent d'un cap que nous avons manqué. « Il nous a également indiqué la méthode pour y parvenir. Elle tient en trois points : dire la vérité travailler avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté ; obtenir des résultats concrets le plus rapidement possible. « Ce cap est clair. Il doit être tenu. Les Français ont, d'ailleurs, dans un souci de cohérence évident, donné au Président et au Gouvernement les moyens de suivre ce cap en désignant une majorité claire et incontestable. Cette majorité claire, nul ne la prend pour un blanc-seing. Elle implique au moins autant de devoirs que de droits. Que le Gouvernement puisse fonder son action sur une majorité forte est une bonne chose. Qu'il ait toujours à l'esprit que l'intérêt général ne se réduit jamais à aucune fraction du peuple français, fût-elle majoritaire, en est une bien meilleure encore. » Quand même ! « Mais la France doit avancer. Il y a, dans ″notre cher et vieux pays″, une envie, une énergie, un espoir qui transcendent les courants politiques. Voilà qui ne devrait surprendre personne les Français nous ont habitués, à travers les âges, à ces sursauts collectifs et à ces retours de confiance, alors même que tout semblait bloqué, voire perdu. En 2017, les Français nous ont dit qu'ils voulaient que la France redevienne enfin elle-même : confiante, courageuse et conquérante. Pour redevenir elle-même, la France doit rétablir la confiance, et d'abord la confiance des Français en l'action publique. Je parle bien de confiance, et pas de morale. Je ne suis pas l'arbitre des élégances et je n'aime pas le mélange des genres. Je ne suis pas non plus un inconditionnel de l'absolue transparence, qui tourne vite au voyeurisme et à l'hypocrisie. Je crois au vieux mot romain de ″vertu″, qui recouvre à la fois l'honnêteté, la rectitude et le courage. Nous avons fait des progrès en la matière depuis près de trente ans, sous la pression souvent, mais de façon très nette. Les règles de financement des partis politiques et des campagnes électorales sont aujourd'hui bien plus strictes et bien plus saines qu'il y a trente ans. Assumons ces progrès. Ils ne comptent pas pour rien. Je veux le dire clairement : nous ne devons jamais laisser discréditer ceux qui ont fait le choix honorable de consacrer une partie de leur vie au service de leurs concitoyens et à la chose publique. Mais, dans leur intérêt même, il faut encore agir, car il y a, à l'évidence, mesdames et messieurs, des pratiques qui ont été longtemps tolérées, mais que le peuple français n'accepte plus. Il s'agit de fixer le cadre qui permettra d'assainir notre vie publique et de rétablir la confiance des Français tout en posant des règles claires pour les élus. C'est l'objet du premier projet de loi qui vous a été soumis. « Comme le Président de la République l'a indiqué hier, nous lancerons également dans l'année les réformes institutionnelles indispensables à la modernisation de notre démocratie. « J'insisterai en particulier sur la réforme de la justice. Dans un État de droit, rien n'est possible sans une justice forte. Si elle est lente, ou lointaine, ou inégalitaire, ou même seulement trop complexe, la confiance se trouve fragilisée. La réforme constitutionnelle renforcera l'indépendance des magistrats. « Dès 2018, une loi quinquennale de programmation des moyens de la justice sera présentée au Parlement. Cette loi permettra à la garde des sceaux d'engager un vaste mouvement de dématérialisation, de simplification et de réorganisation. Avoir confiance dans la justice, c'est pouvoir y recourir simplement et savoir qu'elle tranchera rapidement, en particulier sur les infractions les plus graves lutter contre le terrorisme, la grande criminalité, la fraude organisée, les violences et notamment celles faites aux plus fragiles. Des peines seront renforcées tandis que d'autres incivilités pourront faire l'objet de contraventions plutôt que de procédures plus lourdes mais trop souvent dépourvues d'effet. La construction de 15 000 places supplémentaires de prison est un engagement fort du Président de la République. Il sera tenu, parce que ne pas pouvoir incarcérer ceux qui doivent l'être est inadmissible, mais aussi parce qu'il nous faut traiter dignement les détenus. C'est essentiel pour ne pas transformer les prisons en incubateurs des violences de demain, et c'est essentiel pour nous, car c'est aussi notre dignité qui est en jeu. Nous ferons donc ce qui doit être fait, sans oublier jamais que la prison n'est pas une fin en soi et qu'il est nécessaire d'utiliser l'ensemble des sanctions prévues par le code pénal. Le recours à l'enfermement ne doit pas traduire une paresse de l'esprit qui s'interdirait de réfléchir au sens de la peine, à la nécessité d'empêcher la récidive, à l'obligation de préparer la réinsertion. Rétablir la confiance, c'est aussi rassurer les Français sur le futur de la sécurité sociale. « La sécurité sociale est une partie de nous-même. Elle est, comme le veut une belle formule, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Mais, si tel est le cas, alors traitons-la comme un véritable patrimoine, en l'entretenant, en la préservant, en la rénovant. C'est vrai pour notre système de santé. Les Français y sont attachés, parce que, à juste titre, ils font confiance à leur médecin et aux professionnels de santé, et à l'hôpital, qui reste un pôle d'excellence française. Mais ils constatent que le système est mal coordonné, que la répartition entre urgences et consultations, entre soins de ville et soins hospitaliers n'est pas optimale, que l'on n'évite au fond ni l'exclusion des soins ni l'accroissement des inégalités. « La prévention sera le pivot de la stratégie nationale de santé discutée à l'automne. Des maladies que l'on croyait éradiquées se développent à nouveau sur notre territoire ; des enfants meurent de la rougeole aujourd'hui en France. Dans la patrie de Pasteur, ce n'est pas admissible ! L'an prochain, les vaccins pour la petite enfance qui sont unanimement recommandés par les autorités de santé deviendront obligatoires. En matière de lutte contre le tabac, là encore, il nous faut assumer des choix courageux. Chaque année, le tabac en France entraîne plus de 80 000 décès. C'est la première cause de mortalité évitable, et la consommation quotidienne de tabac augmente chez les adolescents. Ne rien faire est exclu. Nous porterons progressivement le prix du paquet de cigarettes à 10 euros, en luttant sans merci contre les trafics qui minent cette politique de santé autant qu'ils fragilisent ceux qui respectent la loi. Nous créerons un service sanitaire pour les étudiants des filières de santé, afin de leur permettre d'intervenir dans les écoles et les entreprises pour des actions de prévention. Mais prévenir ne suffit pas. Il nous faudra aussi revoir la manière dont est organisé notre système de soins. Nos professionnels de santé sont compétents et dévoués, mais leur action est trop souvent entravée par les rigidités de nos structures, les carcans administratifs, le fonctionnement en silo. Il nous faut donc bâtir des parcours de soins, en favorisant l'interconnexion des professionnels de santé et la circulation de l'information au bénéfice du patient, en mettant en place de nouvelles incitations et de nouveaux modes de rémunération, en mesurant la qualité des soins et en la faisant connaître. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale traduira cette ambition dès cette année. Notre stratégie de santé devra aussi permettre de garantir un égal accès aux soins, pas seulement en droit, mais surtout dans les faits. La ministre de la santé prépare pour le mois de septembre prochain un plan de lutte contre les déserts médicaux, en bonne intelligence avec les collectivités territoriales et les acteurs du monde de la santé. En la matière, la télémédecine offre des opportunités formidables. Nous les favoriserons. « Enfin, notre stratégie de santé devra rompre le cercle vicieux du " renoncement aux soins D'ici à la fin du quinquennat, tous les Français auront accès à des offres sans aucun reste à charge pour les lunettes, les soins dentaires et les aides auditives. Rétablir la confiance, c'est savoir que nous serons tous ici jugés sur la façon dont nous nous comportons avec les plus faibles, pas seulement pour changer le regard que la société porte sur eux, sur le handicap, sur les personnes âgées, sur les plus pauvres, mais aussi pour reconnaître tout ce que nous pouvons recevoir d'eux. Nous revaloriserons dès 2018 l'allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse. Nous simplifierons les procédures pour les titulaires de droits sociaux qui, souvent, par désespoir ou ignorance, ne les réclament plus. Nous renforcerons notre action en matière de lutte contre la pauvreté en insistant particulièrement sur les familles comprenant de jeunes enfants. Ces efforts financiers sont nécessaires. Ils ne sont pas suffisants. « Il nous faut aussi reconnaître et soutenir les solidarités familiales, affectives et financières. Les familles sont de plus en plus diverses, mais leur rôle reste central. La génération de mes grands-parents a été la première à bénéficier de la retraite. La génération de mes parents est la première à bénéficier de la retraite, tout en ayant à assumer une partie de l'aide à ses propres parents. Le changement de civilisation est majeur. Il ne me paraît pas suffisamment pris en compte. La baisse de la natalité, de son côté, réelle depuis deux ans, doit nous alerter.

L'inclusion des personnes en situation de handicap constituera une des priorités du quinquennat. C'est à une mobilisation nationale que j'appelle, sous l'impulsion du Président de la République et sous la conduite de la secrétaire d'État. Les personnes en situation de handicap et celles qui les accompagnent ont droit à la solidarité nationale. Elles ont besoin de bien plus encore, et elles peuvent nous apporter davantage. Un enfant handicapé scolarisé, ce n'est pas seulement une histoire d'argent ou même de justice : c'est une chance pour l'ensemble de ses camarades Une entreprise qui embauche plutôt que de payer une taxe, c'est une communauté de travail plus forte et plus motivée. Les moyens ne pourront pas être illimités. Mais l'énergie que nous y mettrons ne sera pas comptée. « Rétablir la confiance, c'est aussi affermir le lien entre l'État et les territoires. « Nous ne sommes plus à l'époque où la République, encore mal affirmée, n'imaginait son unité qu'au prix de l'uniformité. Les jardins à la française ont leur charme, mais ils se prêtent assez peu au foisonnement d'initiatives dont le pays a besoin et auquel les collectivités sont prêtes. Comme l'a réaffirmé le Président de la République hier, nous voulons donner aux libertés locales toutes leurs forces. » Ah ! « La liberté de s'organiser d'abord, en développant les communes nouvelles ou les regroupements de départements, dès lors que ces fusions ne sont pas contraires à l'intérêt général. La liberté d'exercer ses compétences, ensuite. Osons les expérimentations ! Ne décrétons pas depuis Paris la fin du millefeuille territorial, mais incitons les territoires à adapter localement leur organisation pour tendre, partout où c'est possible, vers deux niveaux seulement d'administration locale en dessous du niveau régional.

En matière de finances locales, nous engagerons avec les collectivités territoriales des discussions indispensables car, si chacun doit bien sûr contribuer à l'effort de redressement de nos comptes publics, cela doit se faire dans le dialogue et le respect, et avec la prévisibilité nécessaire à toute bonne gestion. C'est dans ce cadre que nous engagerons la concertation sur la réforme de la taxe d'habitation, qui doit contribuer, d'ici la fin du quinquennat, à rendre du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Je sais que cette réforme est attendue par les contribuables, mais redoutée par les élus. La taxe d'habitation est aussi nécessaire aux budgets locaux qu'elle est injuste dans son calcul et son évolution pour les contribuables. Améliorer le dispositif pour les collectivités tout en redonnant du pouvoir d'achat pour les citoyens est un objectif qui devrait nous réunir. Rétablir la confiance, c'est aussi éviter de creuser un fossé entre deux France que certains voudraient opposer, mais qui ne peuvent ni vivre ni réussir l'une sans l'autre la France des métropoles mondialisées et la France périphérique. C'est tout l'objectif de la Conférence nationale des territoires, dont la première réunion se tiendra mi-juillet. Nous y proposerons un pacte pour les collectivités, pour les accompagner dans la transition écologique et pour les accompagner dans la transition numérique, en

des hommes ! » Et des femmes ! « Il y a des Français qui n'ont pas de GPS, pas de connectée, dont le téléphone sert à téléphoner, et c'est tout ! Il y a des citoyens qui sont broyés et ignorés par ce monde technique. Le fossé s'agrandit et il n'est pas que générationnel : il est social et parfois géographique. Nos services publics et le monde associatif doivent accompagner ces révolutions numériques. Nous les y aiderons. De même, il y a des votes protestataires qui se sont exprimés en métropole comme en outre-mer ; il faut les entendre. Il y a aussi un vote identitaire, qui s'est notamment exprimé en Corse on peut être, comme je le suis, intransigeant sur les principes républicains sans être, pour autant, ignorant des diversités et des aspirations à la reconnaissance. La France est partout dans le monde grâce à ses outre-mer, sur tous les continents et dans tous les océans du globe. Voilà une richesse, voilà une chance, voilà un défi, Les assises de l'outre-mer seront l'occasion pour l'ensemble du Gouvernement d'être à l'écoute des attentes de chaque territoire et de concevoir ensemble les plans de convergence prévus par la loi pour l'égalité réelle des outre-mer. Pour ce qui concerne l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, cette mandature sera celle de l'aboutissement de l'accord de Nouméa signé il y a vingt ans. S'il n'est pas saisi d'ici mai prochain par le Congrès, le Gouvernement, comme le prévoit la Constitution, organisera la consultation pour l'accession à la souveraineté au plus tard en novembre 2018. L'État jouera pleinement son rôle d'acteur et de garant de ce processus pour conforter le " destin commun " inscrit dans le préambule de l'accord. C'est un engagement personnel que je prends ici, honoré de reprendre le flambeau de Michel Rocard et de quelques autres après lui. La confiance, enfin, c'est tout ce qui nous rassemble. « La France est une nation. Et une nation n'est ni une juxtaposition de territoires ni une addition de communautés, et encore moins une somme d'individus. Une Nation est une adhésion à des valeurs, à une histoire, à une géographie. C'est une culture qui s'assume et se transmet. Être Français, c'est reconnaître des valeurs et partager une culture. C'est reconnaître que la laïcité est une exigence pour la puissance publique, celle de la neutralité absolue à l'égard des cultes. C'est aussi rappeler qu'elle est surtout, pour chacun sur le territoire de la République, une liberté : la liberté de conscience individuelle, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de pratiquer un culte ou de n'en suivre aucun. Le Gouvernement n'acceptera pas que ce principe fondateur soit attaqué, remis en cause ou instrumentalisé. Il le fera respecter sans outrance, en se gardant de provoquer, mais avec une fermeté qui repose sur l'idée simple que la laïcité est, au fond, une condition de ce que nous sommes : la France. Ce qui nous rassemble, c'est aussi la culture. « C'est notre langue, c'est notre patrimoine, c'est ce que nous partageons, c'est ce qui fait que la France est admirée et aimée dans le monde. C'est ce que détestent les porteurs de haine qui, à plusieurs reprises, ont attaqué notre pays. « Et s'ils détestent autant cette culture et ce mode de vie, s'ils haïssent les dessins, les livres, la musique et les spectacles, c'est qu'ils les savent une source inépuisable de réflexion, d'émancipation et de bonheur. Ils savent qu'ils sont libérateurs. Ne nous y trompons pas : la formation dès le plus jeune âge à la culture et à la création rend libre. En les familiarisant avec la longue histoire des arts, en leur en leur faisant découvrir les lieux de culture, en leur apprenant à décrypter l'époque et à découvrir notre héritage, nous élevons l'âme de nos enfants et nous renforçons la cohésion de notre pays. De concert, les ministres de l'éducation nationale et de la culture feront de ce chantier une priorité absolue. « De même, lire rend libre. Plus encore que sous les ors de ses palais, la République vit dans ses bibliothèques. Nous voulons rester, redevenir peut-être, une nation de lecteurs en nous inspirant des initiatives remarquables menées par de nombreuses collectivités territoriales. Accéder aux oeuvres et à la création rend libre. Notre époque bouleverse les modes de diffusion des oeuvres : c'est à la fois une chance et un défi. Profitons-en pour faciliter le plus large accès possible aux biens culturels, avec notamment la création d'un Pass-culture pour les jeunes, comme l'a proposé le Président de la République. Mais ouvrons aussi le débat avec les acteurs géants du numérique dans le cadre européen pour assurer aux artistes les moyens de vivre de leur création et pour participer au financement de cet accès aux oeuvres. Mesdames, messieurs, la France peut renouer avec la confiance. Elle en a, j'en suis certain, les moyens. Elle en a, j'en suis convaincu, l'envie. Elle doit aussi en avoir le courage. Le courage, voilà le deuxième grand axe qui organise le travail du Gouvernement. « Entendons-nous bien. Il ne s'agit pas du courage du Gouvernement, ou de celui de la majorité, ou de celui du Parlement.

Les Français sont courageux. » ! « Ils l'ont été face au terrorisme : pas seulement les policiers, les gendarmes, les militaires ou les douaniers qui luttent contre cette menace et qui en sont trop souvent les cibles, tous les Français Face au danger, ils n'ont pas voulu changer leurs habitudes, encore moins renoncer à leurs valeurs. Il y a dans notre pays une forme de courage tranquille mais réel dont nous pouvons être fiers. La menace est partout, diffuse. Pas un mois ne passe sans que des projets ne soient éventés ou des actes empêchés. Ayons en cet instant une pensée pour les victimes- plus de 200 tués sur notre sol, des centaines de blessés pour leurs proches, qui doivent apprendre à vivre avec la douleur, avec la peine et avec l'absence. « Je veux rendre hommage à tous ceux que nous voyons, policiers, gendarmes, militaires de l'opération Sentinelle, veiller chaque jour sur notre sécurité. À ceux qui combattent sur les théâtres d'opérations extérieures au Sahel ou au Levant. Et à tous ceux que nous ne voyons pas et ne connaîtrons jamais, nos soldats de l'ombre, dont nous pouvons être fiers. Beaucoup sont tombés au service de notre liberté. « Je veux leur dire à tous que nous leur donnerons les moyens de nous défendre. Comme s'y est engagé le Président de la République, une loi de programmation militaire sera adoptée dès 2018. Elle portera l'effort de défense à 2 % du PIB d'ici 2025 et permettra à la France de se battre sur tous les fronts. « Mais je tiens à vous le dire sans détour : il y aura d'autres attaques, d'autres drames, d'autres vies innocentes fauchées. « Nous ne nous y habituerons jamais. Nous ne baisserons pas la garde. À l'image des Français, nous affronterons cette menace avec une calme et froide détermination. « Nous lutterons contre les terroristes avec la plus extrême dureté, sans renier ce que nous sommes : un État de droit et, qui plus est, la République française, une République qui ne peut pas vivre dans un état d'urgence permanent C'est pourquoi le Président de la République nous a demandé de préparer la sortie de l'état d'urgence au plus tard le 1novembre prochain, avec un projet de loi renforçant l'efficacité de notre arsenal législatif contre le terrorisme, sous le contrôle rigoureux du juge. « En parallèle, le ministre de l'intérieur et la garde des sceaux travailleront ensemble pour faire reculer l'insécurité. Au printemps 2018, après des expérimentations, ils porteront ensemble un projet de réforme reposant sur des procédures simplifiées, afin que les forces de sécurité soient libérées de la complexité administrative. Établir une véritable police de sécurité du quotidien, c'est aussi une condition pour rétablir la confiance. Le courage, c'est aussi de regarder en face le défi migratoire. « La pression qui s'exerce aux frontières, dans les Alpes-Maritimes, dans le Calaisis, à Mayotte, en Guyane, qui s'exerce aussi au coeur même du territoire national, comme à Paris, porte de la Chapelle, crée des tensions considérables et lourdes de dangers pour l'ordre public. Cette pression ne faiblira pas : les conflits et l'insécurité économique au Moyen-Orient et en Afrique, les risques liés au climat, les réseaux qui prospèrent en exploitant le malheur et la misère, tout contribue à l'alimenter. Face à cette situation, la France s'est révélée incapable de remplir ses obligations juridiques et morales. « Les demandeurs d'asile relevant effectivement de la convention de Genève attendent l'octroi d'un statut durant de longs mois et dans des conditions parfois honteuses. Les autres, qui sont en réalité des migrants économiques, sont rarement éloignés quand ils sont déboutés. La semaine prochaine, le Gouvernement présentera des mesures qui répondront à trois exigences : une exigence de dignité pour que la France honore sa tradition d'accueil des réfugiés une exigence d'efficacité pour réduire les délais moyens d'instruction des demandes d'asile, de quatorze à six mois, et obtenir l'éloignement effectif des déboutés du droit d'asile une exigence de solidarité et de responsabilité. Avec nos partenaires européens, nous ferons aboutir la réforme du régime européen d'asile commun et mènerons une action en direction des pays d'origine et de transit. « Il s'agit, comme je l'ai dit il y a quelques jours aux préfets que j'ai réunis avec le ministre de l'intérieur, de voir le monde tel qu'il est, sans renoncer à ce que nous sommes. « Accueillir, oui, bien sûr. Aider, oui, évidemment. Subir, non, jamais Le courage, c'est aussi de regarder les choses en face et de préparer l'avenir. « Parlons donc de l'école. « Je suis par mon histoire personnelle un pur " produit " de l'école publique. Deux fois fils de prof, je dois une bonne partie de ce que je suis à mes maîtres, à leur attention, leur persévérance et leur capacité à m'inspirer. Nous connaissons tous le dévouement des enseignants, la passion qui les anime et le rôle qu'ils jouent pour nos enfants. « Et pourtant, toutes les études le démontrent : nous formons " très bien les très bons mais nous creusons les inégalités. Et le niveau moyen de nos élèves n'est pas à la mesure de notre grand pays. « Notre système laisse sortir chaque année encore près de 100 000 jeunes sans qualification. Nous dépensons bien moins que nos voisins dans le primaire, où pourtant tout se joue. Nous dépensons bien plus que les autres pays pour le lycée, notamment parce que notre système est rigide et conçu autour du baccalauréat, que nous conduisons 60 % de bacheliers à l'échec en licence ! « Enfin, scandale absolu, des bacheliers, y compris parmi les plus méritants, se retrouvent exclus par tirage au sort des filières universitaires qu'ils ont choisies

sur les mesures déjà annoncées par le ministre de l'éducation nationale pour l'école et le collège. Elles se concentrent sur l'acquisition des savoirs fondamentaux, le soutien aux élèves et l'autonomie des établissements, et seront en vigueur dès la rentrée prochaine. » Très bien ! « Quant au baccalauréat, nous le ferons profondément évoluer. Une concertation sera lancée dès la rentrée prochaine pour resserrer les épreuves finales autour d'un plus petit nombre de matières et définir ce qui relève du contrôle continu. Nous aboutirons avant septembre 2018 pour une mise en oeuvre complète de cette réforme à compter du bac 2021. Notre ambition est forte aussi pour la filière professionnelle. Le lien entre le lycée professionnel et le monde de l'entreprise, par l'alternance ou par l'apprentissage, doit être resserré. Le lycée professionnel doit aussi être mieux intégré avec les filières post-bac courtes que sont les BTS et les licences professionnelles. Des diplômes de qualification à bac + 1 pourront également être proposés après le baccalauréat professionnel. Nos grandes universités doivent également continuer à se transformer. « Avec l'appui des organismes de recherche, elles doivent continuer à gagner en autonomie, travailler en réseau et se rapprocher du monde économique. C'est dans leurs laboratoires que se construisent l'intelligence collective et la croissance économique de demain. « Les efforts d'investissement ne seront pas relâchés. Nous avons besoin d'universités fortes où formation, recherche et innovation irriguent notre culture et notre économie. Nos universités vont connaître un choc démographique, dont nous devons nous réjouir. Chaque année, ce sont 40 000 étudiants supplémentaires qu'il nous faudra accueillir. Mais nous n'avons pas le droit d'orienter des générations entières vers des formations inadaptées et sans débouchés. Il est temps d'offrir à nos lycéens des " contrats de réussite étudiante qui leur indiquent les prérequis pour réussir dans la filière visée. Nous le ferons dès la rentrée 2018. Il faut aussi garantir un réel droit au retour à l'université tout au long de la carrière, pour compléter et valider en milieu académique les acquis de l'expérience. Notre jeunesse a soif de causes. On n'y répondra pas par des taux de croissance ou par des procédures. La jeunesse veut s'élever. Au siècle dernier, elle a eu trop d'occasions de verser son sang. Le front aujourd'hui est social, environnemental et mondial. Il appelle la mobilisation de la jeunesse, non pour combattre, mais pour construire, partager, déverser le fruit de ses connaissances et de son enthousiasme. C'est aussi pour préparer nos enfants à ce monde qui vient, à cette France que nous voulons grande et belle, juste et forte, que le Gouvernement mettra en place un nouveau service national, conformément aux engagements du Président de la République. La réflexion sur les formes que prendra ce service sera conduite avant la fin de l'année 2017. Le courage, c'est aussi de rénover enfin notre modèle social. Nous sommes, dans notre pays, fortement attachés à l'égalité égalité devant la loi, égalité des droits. Pourtant, nous sentons bien aujourd'hui que cette égalité est malmenée. Le code du travail est le même pour tous, mais le niveau de protection n'est pas le même dans les grands groupes, les PME ou pour celui qui accumule les CDD. Et nous savons aussi que chacun aspire à notre époque à plus de liberté liberté de choisir sa carrière professionnelle, de changer de métier, liberté de créer, liberté d'entreprendre, liberté de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Les catégories traditionnelles qui ont structuré notre vie sociale s'effritent : la frontière entre salariat et travail indépendant, le rôle de la loi et du contrat, la répartition de la valeur. Tout cela est profondément bouleversé par l'impact conjugué de la mondialisation et de la révolution numérique. « Voilà pourquoi nous voulons rénover notre modèle social : pour qu'il crée des protections vraiment efficaces au lieu de les garantir seulement sur le papier ; pour qu'il accompagne celui qui veut prendre un risque, au lieu d'être seulement tourné vers celui qui est déjà installé. « Dès le 6 juin dernier, j'ai défini avec la ministre du travail, et nous avons partagé avec les partenaires sociaux, la feuille de route de cette rénovation sociale. Elle tient en quatre points : renforcer le dialogue social dans l'entreprise et dans les branches ; redonner du pouvoir d'achat aux actifs ; sécuriser les parcours professionnels ; rendre notre système de retraite plus juste et plus lisible. Nous voulons aller vite, car l'urgence sociale est forte. Mais nous avançons sans précipitation. Nous sommes encore dans le temps de la concertation avec les partenaires sociaux

À la fin de l'été viendra le temps de la décision, lorsque les ordonnances seront publiées. « Dès octobre, nous engagerons les chantiers du renforcement de la formation professionnelle, de l'ouverture de l'assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants, de la refonte de l'apprentissage. Nous aurons là aussi de vraies discussions avec les partenaires sociaux et nous présenterons un projet de loi et un plan d'actions au printemps 2018. « Nous appliquerons la même méthode à la rénovation de notre système de retraites, pour le rendre plus juste et plus transparent, pour qu'un euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous. Nous prendrons le temps du diagnostic, de la concertation et de la négociation et nous fixerons le cadre de la réforme à la Entre-temps, nous aurons rendu du pouvoir d'achat aux salariés : la suppression des cotisations salariales sur l'assurance maladie et l'assurance chômage, financée par un transfert sur la CSG, redonnera dès 2018 du pouvoir d'achat à plus de 20 millions d'actifs. » Et les retraites ? ... « Cela représente 250 euros par an au niveau du SMIC. Nous augmenterons aussi la prime d'activité, car le message aux Français est clair : le travail doit payer. « Le courage, c'est enfin de faire face à la vérité sur notre situation financière. Dès ma prise de fonction, j'ai voulu disposer d'une vision nette de la situation de nos comptes publics. Le constat est grave : 8 milliards d'euros de dépenses non financées. Notre dette atteint un niveau insupportable de 2 147 milliards d'euros. Chaque année, la France dépense 42 milliards d'euros pour rembourser ses intérêts. C'est C'est plus que l'intégralité du budget que nous consacrons à notre défense nationale. C'est cinq fois le budget de la justice. Cette dette nous met à la merci des marchés financiers, dont les fluctuations décident de plus en plus de notre avenir. Si une nouvelle crise survenait, nous n'aurions plus de marge de manoeuvre. » Bien sûr ! Nous l'avons dit cent fois ! « Si les taux d'intérêt augmentaient d'un point, et ils augmenteront un jour, c'est l'équivalent du budget de l'enseignement supérieur qui partirait en fumée. Et pourtant, nous continuons à dépenser plus que nos recettes. Je n'aime pas raisonner en pourcentage du PIB : 2,8 %, 3,2 % ... Nous avons anesthésié nos compatriotes à force de parler comme des comptables. La vérité, c'est que quand nos voisins allemands prélèvent 100 euros en impôts et en dépensent 98, nous en prélevons 117 et en dépensons 125. Qui peut penser que la situation est durable ? Mesdames, messieurs, sous le regard inquiet des Français, nous dansons sur un volcan qui gronde de plus en plus fort. Certains continuent pourtant à nier l'évidence. » Pas ici ! « " Combien de fois un homme peut-il tourner la tête en prétendant qu'il ne voit pas ? ", s'interrogerait sans doute le prix Nobel de littérature de l'année 2016 ... « Il y a une addiction française à la dépense publique. Comme toute addiction, elle ne règle rien du problème qu'elle est censée soulager. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer. Mesdames, messieurs, les Français ne croient pas aux solutions simplistes, qu'il s'agisse de la sortie de l'euro ou de l'annulation de la dette. Ils voient bien que tous nos partenaires européens ont fait l'effort de réduire leurs dépenses après la crise financière. Tous, sauf nous. Ils savent qu'il est indigne de demander à leurs enfants de rembourser demain ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se payer aujourd'hui. « Mon objectif est donc de ramener le déficit sous la barre des 3 % dès 2017 et de conduire notre stratégie de finances publiques en fonction de trois règles simples : premièrement, faire baisser la pression fiscale d'un point de PIB sur cinq ans deuxièmement, faire baisser la dépense publique de trois points de PIB sur la même période ; troisièmement, agir en donnant de la visibilité aux acteurs. Je veux d'abord rassurer nos concitoyens : les contribuables ne seront pas la variable d'ajustement du budget ! « Au contraire, les prélèvements obligatoires baisseront de 20 milliards d'euros d'ici à 2022. La France ne peut demeurer la championne à la fois de la dépense publique et des impôts S'agissant de la dépense publique, l'objectif du Gouvernement est ambitieux. C'est de faire en sorte qu'elle soit stable, hors inflation, en 2018 par rapport à 2017 2017 : on ne dépensera pas plus en 2018 qu'en 2017. Tous les autres États l'ont fait, voire ont baissé leurs dépenses. Mais cela n'a été fait qu'une seule fois en France. Encore s'agissait-il de supprimer les mécanismes conjoncturels de soutien qui avaient été institués pendant la crise. Disons la vérité aux Français. » Enfin ! « Pour atteindre ces objectifs sur la dépense publique, il faut agir sur trois leviers. faut stopper l'inflation de la masse salariale du secteur public, qui représente le quart de nos dépenses publiques. « Ensuite, si nous voulons financer nos priorités, et ne pas continuer à paupériser l'État, nous devrons choisir et remettre en cause certaines missions faire bien ce que nous devons faire et arrêter de faire ce que d'autres font mieux que nous. Aucun ministère, aucun opérateur, aucune niche fiscale ne sera sanctuarisé. Partout, nous chasserons la dépense inefficace et le saupoudrage de crédits. de repenser les politiques publiques qui pèsent sur nos actifs sans suffisamment de résultats. Nous dépensons deux fois plus que nos voisins européens dans l'aide au logement

les Français le constatent également dans les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle. « La France est dans les cordes, et aucune esquive ne nous sauvera. J'ai conscience d'appeler à l'effort et au courage. Pour être entendu, il faudra agir de manière juste, transparente et dans la durée, en donnant de la visibilité aux gestionnaires publics et aux Français. « Dès cette semaine, le ministre de l'action et des comptes publics réunira l'ensemble des administrations publiques, pour dessiner une trajectoire et une méthode globale de redressement financier. La conférence des territoires permettra, pour sa part, d'approfondir la concertation avec les collectivités territoriales. « Dès la rentrée, le Gouvernement présentera à la fois le budget 2018 et une loi de programmation des finances publiques qui portera sur toute la durée du quinquennat. « Cette trajectoire devra remettre la sécurité sociale à l'équilibre à l'horizon 2020. Nous devrons d'ici là définir de nouvelles règles permettant de proscrire dans la durée le déficit de nos comptes sociaux. Enfin, nous devrons préserver les équilibres de notre système de retraites, tout en le rendant plus juste et plus lisible. Les nouvelles prévisions du Conseil d'orientation des retraites nous y invitent avec insistance, puisqu'elles indiquent que le retour à l'équilibre, un temps prévu pour 2025, ne pourrait finalement intervenir qu'en 2040. Pour atteindre ces objectifs, nous devons engager une véritable transformation de l'État et de nos services publics. Elle sera progressivement déclinée par ministère

Fixons-nous un objectif simple : avoir des services publics numériques de même qualité que ceux du secteur marchand. Pour ce faire, nous mettrons en place une plateforme numérique et demanderons à chaque administration d'y loger ses applications. Un " compte citoyen en ligne " sera le nouveau lien entre les Français et leurs administrations. Certains diront que c'est trop compliqué, trop ambitieux. J'étais en Estonie la semaine dernière. l'ont fait ... Pourquoi pas nous ? « Cette transformation de l'action passera aussi par une confiance accrue accordée aux fonctionnaires et une modernisation de leur cadre d'action. Je veux leur dire ma fierté de les diriger, mon respect et ma reconnaissance. « Restaurer la confiance, prendre courageusement les décisions que la situation impose, tout cela est nécessaire pour retrouver l'esprit de conquête auquel nous appelle le Président de la République. La France, mesdames, messieurs, doit être de nouveau conquérante. « J'évoquerai tout d'abord le domaine économique. Depuis trop d'années, nous nous résignons à ce que la France tourne au ralenti. Nous nous résignons au chômage de masse. Notre économie ne produit pas assez de revenus, elle ne crée pas assez d'emplois, elle ne donne pas assez de chances à nos enfants. « Au cours des années 2000, nous étions le premier pays d'accueil des investissements étrangers en Europe continentale. Depuis 2010, nous sommes derrière l'Allemagne. En termes d'exportations, nous sommes le seul des grands pays de la zone euro à avoir eu une balance du commerce extérieur déficitaire en 2016, alors qu'elle était bénéficiaire jusqu'au début des années 2000. Surtout, l'économie française croît désormais structurellement moins vite que la moyenne de la zone euro. Cela n'est pas acceptable. Avec les réformes que nous vous proposons, nous voulons redevenir les premiers, en termes d'attractivité, de croissance et de création d'emplois. Une économie attractive, c'est une économie où les charges ne viennent pas freiner le dynamisme de ceux qui créent de la richesse. « Les entreprises doivent retrouver l'envie de s'installer et de se développer sur notre sol plutôt qu'ailleurs. J'annoncerai dans les tout prochains jours, avec la maire de Paris et la présidente de la région d'Île-de-France, des mesures fortes pour améliorer l'attractivité de la place de Paris. Pour favoriser l'embauche, nous baisserons le coût des charges qui pèsent sur le travail, en particulier pour les salaires proches du SMIC. le CICE, sera transformé en allégements de charges, lesquelles seront nulles au niveau du SMIC. La réforme entrera en vigueur au 1janvier 2019. Le taux de l'impôt sur les sociétés sera réduit par étapes de 33,3 % aujourd'hui à 25 % en 2022. » Très bien ! « Il convergera ainsi vers la moyenne européenne. La loi de finances pour 2018 précisera sa trajectoire de baisse, pour donner de la visibilité aux entreprises. « Nous voulons aussi alléger les contraintes qui pèsent sur nos entrepreneurs, en particulier sur les indépendants et les TPE-PME. Des mesures de simplification réglementaire seront prises, et nous engagerons en 2018 la suppression du régime social des indépendants, que nous adosserons au régime général. Une économie conquérante, c'est également une économie qui investit dans l'avenir. Il faut donc réorienter l'épargne des Français vers l'investissement productif. L'impôt de solidarité sur la fortune sera resserré autour du seul patrimoine immobilier, afin d'encourager l'investissement dans la croissance des entreprises. La réforme sera votée dès cette année, dans le cadre de la loi de finances pour 2018, et entrera en vigueur en 2019. La réforme de la fiscalité du patrimoine sera complétée par la mise en place d'un taux de prélèvement unique d'environ 30 % sur les revenus de l'épargne. C'est simple, efficace et compétitif. La France se rapprochera ainsi de la moyenne européenne. « Au bout du compte, vous le voyez, l'ensemble de ces mesures fiscales seront votées dès cette année et engagées dans les deux années qui viennent. Une fiscalité au service de l'activité, c'est important, mais investir dans les secteurs d'avenir est tout aussi décisif. C'est pourquoi nous lancerons un grand plan d'investissement de 50 milliards d'euros dans les domaines de la transition écologique, du développement des compétences, de la santé, des transports, de l'agriculture et de la modernisation de l'État. J'ai missionné Jean Pisani-Ferry pour le concevoir et préparer son déploiement. Une part de cet investissement viendra financer des réformes structurelles de notre économie et de la sphère publique. On économise durablement d'un côté, on investit dans l'avenir de l'autre. Investir dans l'avenir, c'est aussi soutenir notre industrie. Je n'ai jamais été impressionné par ceux qui rêvaient d'une industrie sans usine, et jamais convaincu par ceux qui envisageaient une France sans industrie. « La réalité est sombre. Derrière les succès réels de certains, la désindustrialisation de notre tissu productif s'accélère. Pour redresser la tête et redevenir conquérants, nous devons nous renforcer. Certaines de nos filières, comme l'aéronautique, sont déjà remarquablement intégrées et à la pointe de la technologie, mais nous avons beaucoup d'entreprises industrielles souvent de trop petite taille,

Il nous reviendra aussi de tirer le meilleur parti possible des opportunités ouvertes par la révolution numérique, qui doit être une chance pour tous pour les entrepreneurs qui créent des start-up comme pour les TPE-PME, pour ceux qui sont nés avec la révolution digitale comme pour ceux qui en sont éloignés. La révolution de l'intelligence artificielle est devant nous. Elle est en vérité déjà là. Elle nous touchera tous, dans tous les domaines de la production. Ceux qui font mine de l'ignorer seront les premiers saisis par sa puissance. Nous devons nous y préparer, pour en faire une chance disruptive et non la subir comme une fatalité destructive. Le secrétaire d'État au numérique me proposera dans les trois mois une méthode permettant d'associer les meilleurs spécialistes de ce domaine à la définition d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Renouer avec l'esprit de conquête, c'est aussi relever avec enthousiasme l'incroyable défi que posent les grandes transitions du monde, au premier rang desquelles la transition écologique. Ceux qui, par égoïsme ou inconscience, tournent le dos à l'accord de Paris sur le climat manifestent plus qu'une simple incompréhension du monde qui vient. Ils montrent que, au fond, ils ont peur du futur. L'autruche est sans doute un animal sympathique, mais mettre sa tête dans le sable n'a jamais préparé personne à affronter l'avenir. Il nous revient donc de préparer notre pays et notre planète à cette nouvelle ère, afin de ne pas la subir mais de la façonner. Tout a été écrit sur le sujet, depuis les remarquables livres de Jared Diamond jusqu'aux témoignages saisissants de ceux qui parcourent inlassablement la planète pour éveiller les consciences. Notre rapport aux ressources doit être profondément modifié. Notre cap sera simple à formuler, mais ambitieux et exigeant nous voulons arriver à la neutralité carbone d'ici à 2050. C'est pourquoi nous n'attribuerons plus de nouveaux permis d'exploration d'hydrocarbures. La convergence " diesel-essence " sera atteinte avant la fin de la mandature. » Heureusement ! « La montée en puissance de la fiscalité carbone sera accélérée. Nous diviserons par deux les déchets mis en décharge et recyclerons 100 % des plastiques sur tout le territoire d'ici à 2025. Nous partirons du principe simple qu'il est toujours préférable de taxer la pollution plutôt que le travail, et qu'avant de sanctionner et d'interdire, il vaut mieux encourager et adapter. Le temps des très grandes infrastructures de transport doit céder la place à des politiques tournées vers de nouveaux modes de mobilité qui associent les nouvelles technologies, le secteur public comme le secteur privé, les micro-entreprises comme les champions nationaux. Les assises de la mobilité associeront, dès la rentrée, les usagers, les opérateurs, les collectivités, les ONG, pour orienter les investissements en faveur de déplacements quotidiens plus sûrs, qui désenclavent les territoires. « La loi d'orientation sur la mobilité préparera également l'ouverture à la concurrence, que nous ne devons pas redouter, ni en France ni à l'étranger. Nos opérateurs nationaux de transport sont déjà des champions à l'international. « Autre domaine où une transition profonde s'impose : le logement. Pour construire de nouveaux logements, une loi présentée à l'automne visera à simplifier les procédures, en particulier dans les bassins d'emplois les plus dynamiques. « Les procédures de permis de construire seront accélérées, les recours abusifs sanctionnés. « Au besoin, notamment dans les zones tendues, les autorisations d'urbanisme seront transférées des communes aux intercommunalités pour que les décisions de construire soient prises à l'échelle des bassins de vie. Nous nous fixons aussi dans les dix ans à venir, les passoires thermiques, principales sources de gaspillage énergétique, qui grèvent les budgets des ménages les plus modestes. Être conquérant face aux transformations du monde, voilà bien un principe qui s'applique à l'agriculture.

par l'importance qu'elle occupe dans notre imaginaire et dans notre vie, l'agriculture française a fait bien plus que nourrir, et très bien nourrir, les Français. Elle est aujourd'hui confrontée à de multiples transformations : la pression sur le foncier agricole, la répartition insatisfaisante de la valeur entre producteurs et distributeurs, la concurrence étrangère, la multiplication des normes, la nécessité de préserver l'environnement, la demande croissante de consommateurs pour des productions nouvelles et de qualité. Les agriculteurs français n'ont pas peur de s'adapter. Ils veulent vivre, de leur travail, de leur terre et de leurs compétences. « Les États généraux de

il est inadmissible que des agriculteurs ne puissent se verser un revenu décent et vivent sous le seuil de pauvreté. Ce doit être aussi notre combat pour la politique agricole commune de demain. Ces États généraux devront conforter notre confiance en une alimentation qui réconcilie l'agriculture et l'environnement, en particulier par l'examen sans faux-semblants de la question des pesticides et des perturbateurs endocriniens. « Enfin, vous permettrez à l'ancien maire du Havre que je suis de rappeler que la France conquérante, celle que voulait François I au début de la Renaissance,

Une France conquérante, c'est enfin une France écoutée, respectée et désirée. « Je l'ai dit il y a quelques semaines : la France est de retour, singulièrement en Europe.

ils sont attachés à la construction européenne et à l'euro ; ils veulent une Europe plus concrète, moins tatillonne, plus protectrice. L'agenda européen de ce gouvernement tient en trois idées. « Premièrement, tout faire pour réconcilier les Français avec l'Union européenne.

qu'une politique commerciale de réciprocité, sans naïveté. « Troisièmement, préparer les trois négociations cruciales pour l'avenir de l'Union la redéfinition de notre projet à vingt-sept, avec l'Allemagne et avec ceux de nos partenaires qui voudront aller de l'avant ; la conduite d'une négociation ordonnée de sortie du Royaume-Uni comme préalable au cadre de la relation future les perspectives financières dont dépendra l'avenir des politiques de l'Union après 2020. « Enfin, le Président de la République a rappelé hier que nous ne concevons pas le redressement de notre pays sans une politique internationale qui rende à la France son statut de puissance d'influence mondiale. L'esprit de conquête, c'est aussi nous rendre capables d'attirer à nous l'intelligence de demain, en accueillant toujours plus d'étudiants du monde entier pour enrichir et diffuser nos techniques, notre langue, notre identité c'est attirer toujours plus de richesses grâce à notre offre touristique, qui constitue un atout économique majeur ; c'est montrer au monde qui nous sommes, en organisant de grands événements pendant lesquels la planète nous regardera. La candidature de Paris aux jeux Olympiques de 2024 a mobilisé la France entière autour du sport et de ses valeurs. L'accueil de ces jeux offrira, je l'espère, une chance unique de renforcer la place de Paris au premier rang des grandes métropoles internationales. » Très L'évolution du monde donne toutes ses chances à la France ; ce nouveau monde, en effet, a besoin de science et de raison, d'ordre et de loi, de technologies et de culture, de dialogue et de solidarité. Et la France, c'est tout cela ! « Monsieur le président, mesdames, messieurs, je ne crois pas à l'omnipotence du politique, mais je ne crois certainement pas à son impuissance. Je vous l'ai dit au début de mon propos, et votre assemblée en est la preuve : les bonnes politiques publiques permettent de changer la vie des Français.

Je sais ce que peut la volonté politique lorsqu'elle a le soutien de la représentation nationale et de la majorité du peuple français. J'ai cette volonté. « L'ensemble de l'équipe gouvernementale la partage. Elle travaille avec une méthode, celle de l'efficacité, du dialogue et de la collégialité. Cette méthode de travail, le Gouvernement la propose aux législateurs que vous êtes, en y ajoutant le respect et l'exigence de la vérité. J'ai siégé sur ces bancs, je l'ai dit, et je suis trop attaché au rôle et aux prérogatives du Parlement pour qu'il en aille autrement. OEuvrons ensemble pour que, à la fin de ce quinquennat, la France ait atteint le cap fixé par le Président de la République. Pour que la France ne regrette pas d'avoir choisi l'optimisme et la confiance Travaillons pour que le chômage reflue, pour que les territoires ruraux continuent à vivre, pour que les quartiers libèrent leurs énergies, pour que les expatriés reviennent, que les entrepreneurs innovent, investissent et créent des emplois. Travaillons pour que le mérite soit récompensé. Travaillons pour que nos compatriotes vivent mieux.

Acte est donné de la déclaration de politique générale dont il vient d'être donné lecture au Sénat.

heures trente : Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution.

: « -projet de loi autorisant la ratification de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions

des séances ? ... Ces propositions sont adoptées. Par ailleurs, conformément à l'article 48 de la Constitution et à l'article 29 , alinéas 2 et 3, du règlement, la conférence des présidents a réparti les semaines de séance d'octobre à décembre 2017 entre le Gouvernement et le Sénat- semaines de contrôle et semaines sénatoriales. Le calendrier des semaines de séance sera communiqué

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, si je me présente devant vous dès cette après-midi, quelques minutes seulement après avoir lu la déclaration de politique générale du Premier ministre, Édouard Philippe, c'est parce que le projet de loi inscrit à l'ordre du jour de votre assemblée est d'une importance cruciale, qu'il concerne la sécurité des Français et que, pour le gouvernement auquel j'appartiens, l'on ne saurait transiger avec cette Je veux saluer le président de la commission des lois, M. Philippe Bas, ainsi que le rapporteur du texte, M. Michel Mercier, qui, comme toujours, ont réalisé un excellent travail. également vous remercier d'être présents si nombreux dans cet hémicycle pour l'examen de ce projet de loi important, le premier de ce quinquennat à être discuté en séance publique. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, notre pays vit depuis maintenant deux ans et demi une vague d'attentats terroristes sans précédent dans son histoire. Le bilan est lourd : 239 femmes et hommes ont perdu la vie au cours de huit attaques depuis le mois Plus de 900 personnes ont été touchées dans leur chair ; certaines auront à supporter toute leur vie des séquelles parfois très lourdes. Ce que l'on sait aujourd'hui de cette menace terroriste, c'est qu'elle demeure à un niveau extrêmement élevé. Plusieurs attentats et tentatives d'attentats se sont ainsi produits récemment sur notre sol. Je pense aux deux attaques ayant eu lieu sur les Champs-Élysées, l'une qui, le 20 avril dernier, a coûté la vie à un de nos policiers, et l'autre qui, le 19 juin, visait un escadron de gendarmerie, mais n'a heureusement pas fait d'autres victimes que l'assaillant.

C'est vrai pour l'Allemagne, avec les attaques hivernales du marché de Berlin et de la gare de Düsseldorf. C'est vrai aussi pour le Royaume-Uni, qui a perdu tant de ses enfants dans les attentats de Westminster et, bien sûr, très récemment, de Manchester et de Londres, qui ont ému le monde entier. Les informations dont disposent nos services de renseignement indiquent que le recul de l'emprise de Daech sur les fronts irako-syriens et libyens n'obère pas encore sa capacité à frapper l'Europe et la France. En effet, si les revers subis par l'organisation terroriste n'ont pour l'heure provoqué aucun mouvement massif de retours, grâce notamment aux contrôles opérés à la frontière turque, le risque d'une action conduite par des individus de retour des zones de combat est cependant réel. Par ailleurs, nous avons constaté à l'occasion des derniers passages à l'acte que des individus isolés pouvaient à tout moment connaître une radicalisation rapide et, par des modes opératoires souvent rudimentaires, fomenter des attaques susceptibles d'être extrêmement meurtrières. La menace demeure donc très élevée ; je le constate tous les jours comme ministre de l'intérieur. Pour cette raison, le Président de la République et le Gouvernement n'avaient d'autre choix que de proposer, par le texte que nous étudions aujourd'hui, la prorogation de l'état d'urgence. Vous savez tous dans cette Haute Assemblée quel est le contenu de cet état d'exception, institué par la loi du 3 avril 1955 et modifié voilà tout juste un an par la loi du 21 juillet 2016. Il comporte douze types de mesures. Certaines, comme les perquisitions administratives, les assignations à résidence ou la fermeture par le préfet de lieux de réunion, notamment de lieux de culte, sont bien connues. D'autres le sont moins, mais se sont pourtant révélées très utiles ces derniers mois : je pense à la possibilité d'établir des zones de protection et de sécurité ou de saisir des armes. L'état d'urgence, vous le savez, est en vigueur dans notre pays depuis cette funeste nuit du 13 novembre 2015. Il a été prorogé depuis lors à cinq reprises ; j'ai moi-même eu à voter chacune des prorogations précédentes en tant que membre de cette assemblée. Non parce que nous nous serions tous laissé emporter par une dérive sécuritaire, mais parce que, chaque fois que nous voulions y mettre fin, la situation a exigé que les gouvernements successifs et la représentation nationale le maintiennent, de nouvelles attaques ayant été menées ou pouvant l'être. Durant la campagne électorale, le Président de la République s'était engagé à évaluer à la fois l'intensité de la menace et l'efficacité de l'état d'urgence, avant de prendre une décision sur l'opportunité d'une nouvelle prorogation. J'ai souligné à l'instant combien la menace perdurait. J'en viens au problème de l'efficacité. Permettez-moi de réactualiser quelques données sur le bilan de près de vingt et un mois d'état d'urgence.

des événements comme l'Euro 2016, le Tour de France, les grands festivals que toutes nos régions tiennent en été n'auraient pas pu avoir

À ceux qui penseraient que l'état d'urgence a porté atteinte pendant vingt et un mois à nos libertés, l'organisation de ces événements montre au contraire qu'il a permis de les préserver. Oui, il a permis aux Français de continuer à assister à de grands spectacles, à de grandes manifestations sportives ! Il a permis de vivre, tout simplement. Les possibilités qu'il a en effet offertes aux préfets et au ministre de l'intérieur se sont montrées précieuses pour défendre notre mode de vie, celui que les terroristes entendaient précisément mettre en cause. Autre élément de bilan : les fermetures des lieux de culte dans lesquels sont tenus des propos d'incitation à la commission d'actes terroristes. Depuis la mise en application de l'état d'urgence, fermetures administratives ont été prononcées : seize lieux de culte. Cela peut paraître modeste. Pourtant, il s'agit d'un chiffre important si on le rapporte au nombre de personnes que des prêches fanatiques auraient pu faire basculer dans la radicalisation. Là encore, l'état d'urgence s'est donc révélé d'une réelle utilité, pour éviter que ne grossisse dans notre pays J'en viens maintenant à une disposition qui a suscité de nombreux commentaires : l'assignation à résidence.

préparées, elles sont aujourd'hui utilisées de manière très ciblée et pertinente. Ainsi, à ce jour, 62 personnes seulement se trouvent aujourd'hui en situation d'assignation à résidence 62 personnes, dont les conditions d'assignation sont, grâce aux dispositions prises par les lois du 19 décembre 2016 et du 28 février 2017, ainsi que par la loi du 21 juillet 2016, strictement encadrées, et qui, on ne le rappelle jamais assez, ont la possibilité, parce que nous sommes dans un état de droit, de contester cette mesure devant le juge administratif. Seulement 62 personnes, cela cela dit quelque chose de la manière de la manière dont il fait aujourd'hui usage de l'état d'urgence : de façon adaptée, ciblée et avec une précaution extrême, qui prouve la maturité de notre démocratie. Le dernier point de bilan que je souhaite évoquer concerne les perquisitions administratives. Il s'agit sans doute de la disposition qui a permis d'agir le plus efficacement contre le terrorisme ces derniers mois. Un chiffre suffit à le mesurer : les 4 400 perquisitions menées depuis la mise en vigueur de l'état d'urgence ont permis de saisir 600 armes, dont 78 armes de guerre. Elles ont aussi- mon prédécesseur l'avait rappelé -permis d'éviter de façon directe dix-sept attentats en 2016, auxquels il faut ajouter au moins cinq attentats déjoués depuis le début de l'année. Et je n'évoque même pas le coup d'arrêt qu'elles ont souvent porté à la croissance de certains réseaux et de certaines cellules, dont le développement aurait été à coup sûr porteur de graves dangers pour nos compatriotes. Ces perquisitions se sont donc, la plupart du temps, révélées très efficaces. Et j'ajoute que, comme les assignations à résidence, elles sont désormais conduites de manière extrêmement ciblée, puisque seules 170 perquisitions ont été conduites depuis le 21 décembre 2016, contre 4 376 depuis le début de l'état d'urgence. Cela fait moins d'une par jour sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, messieurs les sénateurs, périmètres de protection, fermeture de lieux de culte, assignations à résidence, perquisitions, vous le constatez, et je crois que les Français en ont pris la mesure,

aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, aux autorités judiciaires et à l'ensemble des services de l'État qui ont veillé à sa bonne mise en oeuvre. Je sais ce que ces vingt et un mois ont supposé pour eux d'engagement sur le plan professionnel de sacrifices sur le plan personnel. Qu'ils soient sûrs que les Français leur en sont reconnaissants, parce qu'ils ont empêché de nombreux attentats attentats et ont très certainement permis de sauver des dizaines, voire des centaines de vies ! Aux adversaires de cet état d'exception, à ceux qui n'ont pas voté pour sa prorogation ou qui voudraient s'opposer à celle que nous proposons, je veux donc dire ceci : imaginez un seul instant que l'état d'urgence n'ait pas été en vigueur ces derniers mois. Imaginez que les forces de sécurité n'aient, par exemple, pas pu perquisitionner à la mi-décembre à Pau. Nous n'aurions pas pu saisir du matériel informatique qui nous a permis d'arrêter et de condamner à de la prison ferme des individus qui, sur leurs messageries cryptées, échangeaient des vidéos morbides et des messages du type : « Tuez-les où que vous soyez ». Imaginez que nos services n'aient pas pu perquisitionner dans les Alpes-Maritimes en avril dernier : nous n'aurions pas pu découvrir qu'une jeune fille de quinze projetait de réaliser un attentat à la bonbonne de gaz dans un bureau de vote. Imaginez que la police n'ait pas pu perquisitionner à Marseille à la fin de décembre 2016 nous n'aurions pas pu saisir au début du mois d'avril ces armes à feu et ces kilos d'explosifs qui étaient destinés à commettre un attentat à l'occasion d'un meeting politique, ni arrêter ceux qui projetaient une telle attaque, telle attaque, laquelle, en cette période, aurait sans doute eu pour conséquence de dresser les Français les uns contre les autres. quand on parle de l'état d'urgence, on ne parle pas seulement de concepts théoriques ! On parle de terroristes arrêtés, d'attentats évités. On parle de vies sauvées. C'est ce que je vous demande d'avoir à l'esprit quand vous vous prononcerez tout à l'heure sur ce projet de loi. Vous avez lu le texte la prorogation que nous vous proposons est de durée modeste, puisqu'elle s'achèvera dans trois mois et demi. Il s'agit aussi de la dernière prorogation que ce gouvernement malgré l'efficacité que je viens de décrire, nous avons, j'ai pleinement conscience que, par définition, l'état d'urgence n'a pas vocation à être permanent. Malgré le contrôle de plus en plus strict dont il fait l'objet, nous avons, j'ai pleinement conscience qu'il provoque des inquiétudes en matière de respect des libertés. C'est pour ces raisons que, à la demande du Président de la République et du Premier ministre, nous avons élaboré avec mes services un scénario de sortie maîtrisée de l'état d'urgence. Ainsi, je porterai dans les jours à venir devant vous un autre projet de loi qui visera au renforcement de la sécurité intérieure. Nous aurons dès demain l'occasion d'en discuter en Son objectif est double : il s'agira de renforcer l'efficacité de notre action en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme, en partant des besoins exprimés par les services, mais avec la volonté de limiter strictement les mesures nouvelles à la seule lutte contre le terrorisme, dans des conditions beaucoup plus ciblées qu'en période d'état d'urgence, en apportant ainsi le maximum de garantie quant à la préservation de nos libertés individuelles et collectives. Notre obsession, et je sais qu'elle est partagée sur ces travées, est toujours la même : protéger les Français.

-ne comprendrait que, face à un ennemi n'admettant aucune autre règle que celle de la haine et la barbarie, notre pays se désarme de manière unilatérale. Mesdames, messieurs les sénateurs, en filigrane des controverses qui accompagnent ce projet de loi, il y a un débat que nous connaissons bien dans cet hémicycle : le débat entre sécurité et liberté, avec cette idée, développée par certains, qu'assurer une sécurité accrue ne pourrait se faire qu'au détriment des libertés. Je crois pour ma part qu'une telle opposition relève de l'aporie et que, au contraire, sécurité et liberté sont deux valeurs intimement liées ; l'une ne va pas sans l'autre. effet, je l'ai dit, il faut pouvoir assurer un climat de sécurité pour que les Français soient au quotidien en mesure de sortir de chez eux, de se rendre à un événement sportif et culturel, tout simplement Comme il faut pouvoir assurer un climat de sécurité pour permettre à chaque Français d'envisager l'avenir avec confiance, de se projeter, de se construire. On l'oublie souvent, mais l'un de nos textes fondateurs, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, indique ce lien organique entre sécurité et liberté, puisque, en son article II, il inscrit dans une même phrase liberté et sûreté.

d'augmenter la durée de l'assignation à résidence, puisqu'il faut prouver qu'il existe un moyen nouveau ou des circonstances nouvelles attestant que

Triste record, lorsque l'on sait que l'état d'urgence est un état d'exception, dangereux pour l'État de droit, puisqu'il permet de déroger à certaines garanties et libertés fondamentales. C'est pourquoi son entrée en vigueur n'est permise par le droit international que sous certaines conditions bien précises la Nation doit être en danger ou faire face à un péril imminent d'une extrême gravité. Or il semblerait, selon le gouvernement de M. Philippe, que la nation française soit entrée dans un état de danger constant, alors que de nombreux responsables alors que de nombreux responsables de la lutte antiterroriste eux-mêmes conviennent que l'état d'urgence n'a été nécessaire que durant quelques semaines après les attentats de novembre 2015. mes chers collègues, le Premier ministre et le Président de la République- ce dernier l'a clairement rappelé hier -nous mettent « en marche » pour un état d'urgence permanent, à l'ère de la suspicion généralisée, non seulement avec cette nouvelle prolongation

que le caractère disproportionné et attentatoire aux libertés publiques des dispositions d'exception qui le composent n'a cessé d'être démontré par de nombreux syndicats, associations, organismes de défense des droits de l'homme ou autres universitaires et professionnels du droit. Assignations à résidence, perquisitions administratives, contrôles d'identité et fouilles de véhicules, placement sous bracelet électronique de toute personne suspecte : toutes ces mesures viennent éclabousser libertés publiques et séparation des pouvoirs, en passant sous le contrôle des préfets et du ministère de l'intérieur, sans efficacité avérée Un glissement dangereux est en passe d'être entériné avec ce projet de loi : les stratégies de maintien de l'ordre viennent rogner nos droits fondamentaux afin de prévenir des risques potentiels. La justice par la preuve objective est est peu à peu bafouée, laissant place à une justice du soupçon, comme le confirment de nombreux juristes, à l'instar de Mireille Delmas-Marty, professeur honoraire au Collège de France. Alors que, outre-Manche, Mme Theresa May s'enferre, elle aussi, dans une logique sécuritaire plus que préoccupante, à la suite des terribles attentats de Manchester et de Londres, considérant les droits de l'homme comme des obstacles à la lutte contre le terrorisme, les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen appellent l'exécutif de notre pays à se ressaisir. Ces logiques servent précisément celles qu'elles prétendent combattre, notamment l'asservissement par la peur que les terroristes veulent instiller en chacun de nous en s'attaquant aux droits fondamentaux, piliers de nos démocraties. Les dérives de l'état d'urgence ont en effet été constatées à maintes reprises. Des mesures fondées sur l'état d'urgence ont été prises en de nombreuses occasions dans le cadre général du maintien de l'ordre, sans aucun lien avec la menace terroriste. Elles ont servi en particulier à restreindre le droit de manifester de la COP21 aux mobilisations contre la loi travail, l'état d'urgence a permis d'interdire au moins 155 manifestations et d'empêcher des centaines de personnes de manifester par des assignations à résidence et des interdictions individuelles de manifester, sans que ces personnes aient aucun lien avec la menace terroriste. Les interdictions sont prises sur des motifs souvent extrêmement flous et vagues. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 juin 2017, a déclaré le 3° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence contraire à la Constitution, arguant que cette mesure avait été prononcée sans qu'elle soit justifiée par la prévention d'une atteinte à l'ordre public. le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et venir et le droit de mener une vie familiale normale ». Nous défendrons tout à l'heure un amendement visant à réellement prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel, considérant que la réécriture proposée par le Gouvernement et par le rapporteur en commission n'est pas satisfaisante et reprend, malgré les prétendues garanties introduites, l'interdiction de séjour. Et si, depuis le début de l'année, l'emploi de cette interdiction de manifester, qui se révèle anticonstitutionnelle, a diminué, il y a fort à craindre une recrudescence de son usage à la rentrée, avec la réforme du code du travail par ordonnances. Néfaste pour notre démocratie, ce genre de disposition vient également alimenter une fracture sociale dangereusement renforcée par l'état d'urgence. En effet, les personnes perquisitionnées et assignées à résidence de manière manifestement injustifiée et abusive ont alors vécu une dégradation des relations avec leur voisinage et parfois avec leur entourage direct. La conséquence est inévitable : sentiment d'être mis à l'écart, d'être des citoyens de seconde zone. En quelque sorte,

vous l'aggravez brutalement et répondez ainsi à l'urgence patronale ! Les projets de loi que M. Macron nous soumet pour entamer son mandat viennent faire écran par rapport à l'urgence qu'il y a à combattre la casse du code du travail, qui sera parachevée en parallèle. Toutefois, nous ne sommes pas dupes, et tant que nos sièges, tout à gauche, seront pourvus, vous nous entendrez dénoncer vos savantes manoeuvres ! Finalement, vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe communiste républicain et citoyen votera unanimement contre cette énième prorogation de l'état d'urgence.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, la sixième prorogation de l'état d'urgence que nous examinons aujourd'hui a été étudiée par le Conseil d'État et déposée sur le bureau de notre assemblée conjointement à un projet de loi relatif à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme, ce qui n'est pas anecdotique. En agissant de la sorte, le Gouvernement entend donner des gages pour une sortie rapide de ce régime exceptionnel. Nous discuterons précisément de ces prochaines réformes le moment venu. Pour l'heure, la question porte uniquement sur l'opportunité de proroger l'application du texte du 3 avril 1955, du 15 juillet 2017 au 1 novembre 2017. Mes chers collègues, vous le savez, la défense des libertés est l'une des valeurs cardinales de notre groupe. Nous avons donc été particulièrement attentifs aux réserves formulées par le vice-président du Conseil d'État lors de sa précédente prorogation, ainsi qu'aux craintes exprimées par les associations de défense des droits de l'homme. De la même manière, la répétition de ces prorogations ne doit pas nous conduire à traiter une telle mesure comme une formalité. Sur ce point, notre vigilance est toujours entière. L'histoire nous enseigne que l'équilibre entre sécurité et liberté n'est pas intangible, qu'il s'adapte à l'évolution des circonstances temporelles. L'installation d'une menace terroriste permanente constitue évidemment un élément de nature à bouleverser ce rapport entre libertés et sécurité. S'il est difficile de mesurer depuis les travées du Parlement l'imminence d'attaques potentielles- nous nous en remettons sur ce point totalement aux rapports des services de renseignement -, il est nécessaire en revanche de prendre acte de l'évolution de la perception sécuritaire de nos concitoyens. Toute perception, même excessive, est un fait politique à prendre en compte. Face à cette nouvelle perception, la précédente législature n'est pas restée inactive, au contraire ! Au-delà des prorogations de l'état d'urgence, cinq lois relatives à la lutte contre le terrorisme ont été adoptées. Un nouveau régime d'utilisation des armes à feu pour les forces de l'ordre a été instauré, des procédures dérogatoires ont été instituées, le recours à des technologies a été autorisé avec son lot de risques pour le respect de nos vies privées. Enfin, de nouvelles incriminations ont été insérées dans le code pénal. Votre prédécesseur, monsieur le ministre d'État, a également obtenu d'importantes avancées au niveau européen, avec la conclusion des accords sur le PNR, le, et sur l'harmonisation des règles de neutralisation d'armes à feu. Nous vous souhaitons de poursuivre sur cette ligne ! Beaucoup Beaucoup a donc déjà été fait pour doter notre pays des moyens de se protéger hors du régime exceptionnel de l'état d'urgence, bien qu'il reste encore des sujets de préoccupation ; la prolifération des armes à feu sur notre sol en est un, qui mériterait que l'on y consacre un Grenelle dans le contexte actuel, alors que les terroristes ne désarment pas en Europe et que le Gouvernement entre en fonction, il est nécessaire de lui permettre de commencer à agir dans des conditions sereines. C'est pourquoi, dans le souci constant d'apporter notre soutien aux forces de l'ordre, qui pourraient souffrir les premières d'un flottement législatif, le groupe du RDSE est en majorité favorable à cette nouvelle prorogation. En attendant la nouvelle feuille de route antiterroriste, les contrôles effectués par le juge administratif et le Conseil constitutionnel sont suffisants pour protéger nos libertés, au regard des circonstances particulières que j'évoquais. L'existence de décisions d'annulation ou de censure prouve à elle seule la vitalité de ces contrôles. En conclusion, nous espérons que l'adoption de cette prochaine loi de sécurité intérieure nous permettra de sortir du paradoxe d'un état d'urgence devenu permanent, pour passer au temps de l'application. « Il n'est pas toujours nécessaire de faire des lois, mais il l'est toujours de faire exécuter celles qui ont été faites » écrivait au XVII siècle le philosophe empirique anglais John Locke. Nous avons tous ici conscience que nous ne parviendrons pas à écrire une loi qui garantisse un risque terroriste zéro. Ne tombons pas dans le piège de l'immobilisme que nous tendent les djihadistes. Dans le respect de la liberté du vote qui est le fondement du groupe du RDSE, ses membres se prononceront en faveur de la prorogation, à l'exception de deux votes contre, pour les réserves que j'ai énoncées.

Je ne prétends pas qu'il ne doit jamais plus être mis en oeuvre si des circonstances dramatiques devaient à nouveau l'exiger, mais la prolongation sans fin, chacun le sait, pose plus de questions qu'elle ne résout de problèmes. Nous ne pouvons pas vivre en permanence dans un régime d'exception. Il faut donc revenir au droit commun, tel qu'il a été renforcé par le législateur, et agir avec les bons instruments. Nous avons tout l'appareil législatif permettant de répondre dans la durée à la situation qui est la nôtre.

Ce n'est pas en changeant les mots que l'on changera les choses et les règles en vigueur ! Nous aurons donc un grand débat sur l'État de droit, sur l'équilibre à trouver entre

mais le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement, est censé le contrôler : « L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est en effet la sixième fois que nous délibérons sur la prolongation de l'état d'urgence. Nous le faisons scrupuleusement, comme nous l'avons toujours fait.

impérieuse et pour des motifs de péril imminent. L'actualité récente comme les terribles attentats si meurtriers

en prorogeant une nouvelle fois l'état d'urgence, ne court donc guère le risque d'être censuré par le Conseil constitutionnel, si d'aventure celui-ci était saisi. Pourtant, il est vrai que vivre sous le régime de l'état d'urgence depuis le mois de décembre 2015, c'est-à-dire depuis près de deux ans, soulève un certain nombre de questions quant à la durée de mise en oeuvre de ces pouvoirs exceptionnels. Ces questions n'auraient pas l'intensité qu'elles sont en train de prendre

qu'un certain nombre d'assignations à résidence avaient permis d'améliorer la surveillance d'individus, lesquels ont pu ensuite être traduits devant la justice. Mais, au fur et à mesure que nous vivons dans cet état d'urgence, nous constatons qu'il y a moins d'assignations à résidence et que les perquisitions sont moins fécondes. Ce n'est pas surprenant, car les malfaiteurs qui savent que l'on peut perquisitionner de nuit comme de jour, sans la demande du juge, ont pris toutes les précautions nécessaires pour dissimuler les objets qui révéleraient leurs intentions criminelles. Quant aux assignations à résidence, certaines durent depuis deux ans,

traduction devant la justice des individus concernés est-elle réellement utile ? N'oublions pas que nous disposons, par ailleurs, de moyens de surveillance particulièrement étendus depuis l'adoption de la loi sur le renseignement.

qui inspire cette forme de pédagogie consistant à dire aux Français : « Rassurez-vous, nous ne lèverons l'état d'urgence qu'après avoir durci l'état de droit ordinaire ».

dans le droit commun de très nombreuses mesures. Nous sommes bien placés pour en parler, parce que l'initiative est très souvent venue du Sénat.

un projet de loi visant à renforcer la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Nous ne l'avons pas attendu : dès le mois de décembre, nous étions prêts et nous avons déposé notre proposition de loi, laquelle a été adoptée par le Sénat le 2 février 2016. Cela n'a pas empêché le Gouvernement de poursuivre sa tâche, nous faisant d'ailleurs prendre, au passage, encore un peu de retard

par la police, par le parquet et par les juges pour prévenir, combattre et réprimer le terrorisme. Nous avons été encore plus dans la loi du 21 juillet 2016, consécutive aux attentats de Nice, qui renouvelait l'état d'urgence, et qui, de surcroît,

pour les terroristes. Nous avons multiplié les incriminations permettant de poursuivre un individu qui consulterait régulièrement des sites incitant à la commission d'attentats terroristes. Nous avons permis que soient poursuivis des individus qui reviennent de camps d'entraînement djihadistes.

permettant de lutter contre le terrorisme, nous sommes à votre écoute. Je pense, pour ma part, que le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme dans les périodes suraiguës que nous avons connues, c'est encore l'état d'urgence. Il présente en effet des avantages. Le premier est le contrôle du Parlement. Nous avons ainsi mis en place un comité de suivi au sein de la commission des lois, que je préside, dont Michel Mercier est le rapporteur spécial. La commission des lois a été dotée à plusieurs reprises des pouvoirs d'une commission d'enquête, et nous avons prévu dans la loi que vous devez nous informer de chaque décision que vous prenez. Nous avons la possibilité d'utiliser nos pouvoirs d'investigation. Enfin, les pouvoirs exceptionnels n'étant conférés que pour une durée déterminée, vous êtes obligés de venir nous rendre compte, ce qui est une garantie importante pour les Français. Qui plus est, jamais on n'aura vu autant de décisions du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel

de l'arsenal juridique autorisé par l'état d'urgence, sans pour autant aller jusqu'à dénaturer un certain nombre de règles fondamentales qui nous permettent de respecter

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, madame la ministre, mes chers collègues, si le sujet- la sécurité des Français - n'était pas aussi grave, j'utiliserais volontiers le fameux proverbe : « Faute de grives, on mange des merles ». En effet, faute de mettre en place un contrôle strict et systématique à toutes nos frontières pour savoir qui entre sur notre sol, vous nous faites proroger l'état d'urgence. Faute d'expulser les étrangers fichés S connus pour leurs liens avec des organisations terroristes, vous nous faites proroger l'état d'urgence. Faute d'appliquer l'article 411 du code pénal à l'encontre de nos compatriotes dont il est avéré qu'ils ont des liens avec des organisations terroristes, vous nous faites proroger l'état d'urgence. Faute de restaurer l'État de droit dans tous les quartiers de notre territoire et de mettre en place un vaste plan de désarmement des banlieues, vous nous faites proroger l'état d'urgence. Faute de fermer la centaine de mosquées dans lesquelles on prêche la haine de nos valeurs et la haine de la France, vous nous faites proroger l'état d'urgence. Faute d'expulser les imams étrangers dont les propos poussent certains à rejoindre le camp des islamistes radicaux, vous nous faites proroger l'état d'urgence. Faute d'une politique étrangère claire, qui doit réduire au strict minimum les échanges avec les pays soupçonnés de soutien au terrorisme, faute de pouvoir renforcer les moyens humains et techniques des services de renseignement mis à mal par les deux quinquennats précédents, en raison d'une soumission totale à l'austérité imposée par l'Union faute de mettre en place une politique pénale ferme, rapide et financée, faute de limiter drastiquement l'immigration, dont les liens avec l'islamisme radical sont bien avérés, quoi qu'en disent les chantres du politiquement correct, vous nous faites proroger l'état d'urgence. Bref, faute de présenter une politique ambitieuse en matière de sécurité, vous nous faites proroger une énième fois l'état d'urgence ! Nous allons voter ce texte, car c'est mieux que rien, mais nous le voterons en n'oubliant pas que cet état d'urgence n'a pas empêché l'attentat islamiste de Nice, il y a presque un an, l'assassinat du père Hamel, les attaques sur les Champs-Élysées, dont l'une fut fatale à Xavier Jugelé, l'attaque contre des policiers sur le parvis de Notre-Dame, de Notre-Dame, l'attaque contre un agriculteur dans le Tarn ou encore l'assassinat de Sarah Halimi, pour ne reprendre que les actions des islamistes depuis un an ! Votre idéologie vous aveugle, et vous empêche de prendre les mesures les plus efficaces pour protéger les Français. Ainsi, vous vous obstinez à faire voter l'état d'urgence, alors que l'application stricte de nos textes et un retour de notre pleine et entière souveraineté permettraient déjà, nous en sommes convaincus, de protéger plus efficacement les Français, même si, bien évidemment, nous savons que le risque zéro n'existe pas ! Je conclus mon propos en rendant un hommage appuyé aux forces de l'ordre, aux militaires et aux différents services de renseignement qui, avec courage, abnégation et dévouement, travaillent durement à la protection de notre pays et de nos compatriotes ! Monsieur le ministre d'État, contrairement à ce que disait votre prédécesseur, nous ne voulons pas nous habituer à vivre avec le terrorisme islamiste

qui continue à peser sur notre pays et sur chacun de nos concitoyens. Nous devons donc faire l'effort d'accumuler le maximum d'outils de précaution et de prévention. C'est à cela que sert l'état d'urgence. Au moment où le Gouvernement nous demande une dernière prolongation pour les trois prochains mois, ayons en mémoire les réflexions et les constats que nous avions faits non seulement lors de nos débats,

Mais qui nous dit qu'une bonne partie de la détection des risques, d'embryons de réseaux et de préparatifs d'actes terroristes n'ont pas été découverts à partir de la chaîne de renseignement déclenchée par certaines de ces perquisitions ?

comme des pivots, des organisateurs de réseaux, il est tout de même plus simple de les avoir à l'oeil dans un espace géographique déterminé que d'engager des dizaines de fonctionnaires de police qualifiés pour

beaucoup de prudence et d'ouverture, sans fermer aucune porte, relatif au projet de loi antiterroriste sur lequel nous allons délibérer dans quelques jours. Je tiens à apporter le soutien déterminé de notre groupe au Gouvernement sur cette dernière prolongation. Il est nécessaire, bien sûr, que ces mesures administratives et celles qui leur succéderont soient entourées par un ensemble plus vaste : les mesures de déradicalisation et le renforcement du renseignement, en particulier de la capacité d'analyse. En réaffirmant

pour la sixième fois depuis le 20 novembre 2015, nous voici réunis afin d'examiner une demande de prorogation de l'état d'urgence. La dernière fois que nous avons évoqué cette question dans l'hémicycle, c'était en décembre dernier. Depuis cette date, nous avons de nouveau été frappés par le terrorisme. Récemment, à deux reprises et en plein coeur de Paris, des policiers ont encore été pris pour cible par des individus armés. Xavier Jugelé l'a payé de sa vie. Nos voisins européens n'ont pas été épargnés : Berlin, Londres, Manchester, Saint-Pétersbourg ou encore Stockholm ont récemment été victimes de cette barbarie. Malgré tout, cette nouvelle prolongation pourrait légitimement susciter des interrogations. Chacun sait ici qu'au cours des derniers mois nous avons déjà modifié un certain nombre de dispositions de droit commun renforçant sensiblement les moyens de la lutte antiterroriste afin de préparer une sortie de l'état d'urgence. Cette perspective de sortie est d'ailleurs évoquée par le Conseil d'État dans chacun des avis qu'il a rendus depuis la première prorogation. Comme le Conseil, plusieurs d'entre nous ont remarqué, à juste titre, que l'état d'urgence n'avait pas vocation à être prolongé indéfiniment. Nous devons conserver à l'esprit cet impératif. Mais la question la plus fondamentale, qui doit rester notre préoccupation immédiate, est la sécurité de nos concitoyens : l'état d'urgence est-il toujours justifié, étant donné le niveau de menace pesant sur le France ? Les moyens donnés par l'état d'urgence sont-ils toujours indispensables ? Notre groupe, dans son ensemble, est convenu que la prévention mais aussi la résilience face au terrorisme sont plus que jamais d'actualité. Au regard de la persistance durable de la menace terroriste à un niveau très élevé sur notre territoire, la prolongation de l'état d'urgence s'avère être nécessaire. Mais cette sixième prorogation doit être la dernière. Le Président de la République l'a solennellement annoncé à Versailles ; nous espérons que cet engagement pourra être et sera tenu. Des éléments figurant dans l'exposé des motifs du projet de loi que nous examinerons cet été nous incitent à le penser. Plusieurs mesures permanentes prévues dans ce texte renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme visent ainsi à prévenir de manière plus efficace les actes de terrorisme et devraient permettre- nous l'espérons très fort -« une sortie maîtrisée de l'état d'urgence Par ailleurs, ce projet de loi est utile : il nous offre la possibilité de tirer les conséquences de la décision QPC du 9 juin 2017 du Conseil constitutionnel, par laquelle ce dernier a déclaré contraires à la Constitution les dispositions relatives à l'interdiction de séjour de la loi de 1955. L'amendement du Gouvernement, adopté en commission, vise à rétablir la possibilité pour les préfets de prendre des mesures d'interdiction de séjour en respectant les prescriptions du Conseil constitutionnel. Sans cette modification, l'interdiction de séjour dans le cadre de l'état d'urgence aurait été abrogée le 15 juillet 2017, ce que nous ne pouvions bien évidemment nous permettre.

Cela fait presque deux ans maintenant que son analyse et sa parfaite connaissance du sujet nous permettent de voter de manière éclairée- du moins nous l'espérons fort. Nous devons à nos concitoyens un discours de vérité : non, l'état d'urgence ne permet pas d'éviter les attentats et nous en avons eu la terrible démonstration au cours de ces derniers mois. Non, l'état d'urgence n'est pas suffisant pour faire face à cette menace sans précédent. Pour autant, il demeure aujourd'hui absolument nécessaire. Cela ne doit pas nous faire perdre de vue que la voie judiciaire est l'outil premier et incontournable de la lutte antiterroriste et que, très vite, c'est dans un système hors urgence, pérenne, que notre pays devra s'inscrire et s'adapter à la menace. Nous ne gagnerons la guerre contre le terrorisme qu'en réformant la justice, en préservant et en respectant les libertés individuelles, et donc aussi, comme l'a souligné hier le Président de la République, les juridictions de l'ordre judiciaire. Nous ne gagnerons la guerre contre le terrorisme qu'en poursuivant et en accroissant au niveau européen, comme le fait déjà avec force Eurojust, une coordination étroite de nos systèmes d'information.

Lorsqu'on est ministre de l'intérieur, il y a un avant et un après. Vient le moment où l'on commence à connaître

Je n'ai jamais été de ceux qui pensaient qu'il y avait un « avant » et un « après » qui changeait radicalement.

que le Sénat a été, sur ces problématiques, particulièrement à l'oeuvre, en apportant de la matière à la réflexion du Gouvernement. Je ne doute pas qu'il continuera à le faire

qui vise à supprimer la possibilité de recourir aux perquisitions administratives. Je veux dire à mon collègue et ami Jean-Yves Leconte que je ne comprends pas les deux motivations qu'il met en avant. Premier

pose plus de questions qu'elle ne résout de problèmes. Nous ne pouvons pas vivre en permanence dans un régime d'exception. Il faut donc revenir au droit commun, tel qu'il a été renforcé par le législateur et agir avec les bons instruments. Nous avons tout l'appareil législatif permettant de répondre, dans la durée, à la situation qui est la nôtre. » J'ai cité le candidat Emmanuel Macron dans son livre-programme. Le candidat devenu Président de la République aurait-il oublié ces propos si raisonnables ? On nous demande à nouveau de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 1 novembre prochain, le temps de faire adopter une nouvelle loi qui va institutionnaliser ce régime d'exception. Pourquoi d'autres pays européens cibles du terrorisme, comme la Belgique, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, n'ont-ils pas eu recours à l'état d'urgence ? Leur vision de la démocratie ne fait probablement pas fi des libertés individuelles que l'état d'urgence met en cause. Ajoutons que l'état d'urgence en France n'a pas évité la tuerie de Magnanville, ni celles de Nice, de Saint-Étienne-du-Rouvray, des Champs-Élysées, encore. Actuellement, il sert surtout à couvrir nos dirigeants au cas où il y aurait un attentat. Il permet aussi ce que l'on appelle avec beaucoup de pudeur « le maintien de l'ordre Les chiffres fournis en décembre 2016 par le ministère de l'intérieur font état de 4 292 perquisitions, de 612 assignations à résidence, dont aucune pour des faits liés au terrorisme. selon un rapport d'Amnesty International, tous les trois jours environ, une manifestation est interdite en France sous ce prétexte. Une fois de plus, sans trembler, je voterai donc contre l'état d'urgence. Personne ne